J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2018 et sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas parvenues à l'adoption de textes communs. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème : « Le retour des djihadistes en France », organisé à la demande du groupe La République En Marche. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

déradicalisation, prévention, réponse judiciaire et carcérale, la lutte contre le djihadisme et ses conséquences est l'un des grands défis qui se posent actuellement en France et, plus largement, en Europe. Il n'y a pas de solutions simples pour le relever. Il nous faut avoir sur cette question un débat constructif, qui réunisse toutes les compétences, tous les savoirs et toutes les intelligences. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Vous le savez, le phénomène djihadiste n'est pas nouveau. En effet, l'émergence de la mouvance djihadiste trouve son origine dans l'invasion soviétique de l'Afghanistan et le conflit qui s'ensuivit, à partir de 1979. Des combattants afghans, les moudjahidines, mènent le combat contre l'URSS au nom du djihad et de la défense de l'islam. L'Afghanistan attire alors plusieurs dizaines de milliers de combattants étrangers issus de l'ensemble du monde musulman, en particulier des pays arabes. À la fin de la guerre, en 1989, ces combattants étrangers cherchent à rentrer dans leurs pays d'origine ou à rejoindre d'autres théâtres, afin de propager leur idéologie. Ces « vétérans afghans » vont jouer un rôle majeur dans la création et le développement de groupuscules djihadistes à travers le monde, en particulier dans les pays arabes et en Asie, mais aussi en Europe. Au cours des années quatre-vingt-dix, le conflit en Bosnie et la « décennie noire » en Algérie contribuent à l'internationalisation de la mouvance djihadiste et à son développement sur le territoire européen. Plusieurs milliers de combattants étrangers, dont de très nombreux Européens, partent combattre dans les Balkans. À leur retour, certains forment des cellules djihadistes en Europe. Le conflit algérien est à l'origine de la première grande vague d'attentats djihadistes en France et en Europe. La fin des années quatre-vingt-dix et le début des années 2000 sont marqués par la montée en puissance d'Al-Qaïda, qui culmine avec les attentats du 11 septembre 2001. L'émergence de Daech en Syrie et en Irak, à partir de 2006, marquée par la proclamation du « califat » au mois de juin 2014, constitue un bouleversement majeur pour la scène djihadiste internationale. En effet, le d'Al-Qaïda est remis en cause. Sur le plan idéologique, la spécificité de Daech réside dans son projet étatique de fondation d'un califat islamique, fondé sur la maîtrise de territoires en Syrie et en Irak. Ce projet est en rupture avec la doctrine d'Al-Qaïda, qui prône un djihad déterritorialisé, centré sur la lutte contre l'ennemi lointain. Impressionnés par les succès initiaux de Daech en Syrie et en Irak, plusieurs dizaines de groupes djihadistes font allégeance à l'organisation. Ils en reprennent le discours, les symboles et les méthodes. Pour sa part, Daech a annoncé la création de plusieurs « wilayas », c'est-à-dire provinces, censées symboliser l'expansion du prétendu califat, en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Afrique de l'Ouest, dans le Caucase ... L'émergence de Daech s'est aussi traduite par une transformation et une intensification de la menace. Daech incite à la haine à travers sa propagande sur internet et sur les réseaux sociaux, favorisant le passage à l'acte d'individus radicalisés. Ce phénomène de « loup solitaire » est nouveau et donc très difficile à appréhender. Là aussi, notre débat de ce soir doit être éclairant. La plupart des jeunes radicalisés ont eu des démêlés avec la justice, affichent un passé de délinquant et ont commis des vols ou fait du trafic. La grande majorité a vécu des périodes d'emprisonnement plus ou moins longues. Pratiquement tous n'avaient pas de pratiques religieuses et sont devenus musulmans ou convertis djihadistes sous l'influence d'un gourou, de copains, à partir de leurs lectures sur internet ou en prison. Enfin, la grande majorité a fait le voyage initiatique dans un pays du Moyen-Orient ou des zones de guerre : l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan L'utopie régressive de la néo-Oumma- la communauté des musulmans au-delà de leur nationalité -, combinée au rôle du preux chevalier du djihad, exerce une indéniable fascination non seulement sur certains jeunes des banlieues, mais aussi, pour des raisons différentes, sur des jeunes de la classe moyenne en quête de sens qui constituent le second groupe « amoureux » du djihadisme depuis la guerre civile en Syrie en 2013. Pourtant, il est important de retenir que ces jeunes ne sont au départ ni pieux ni radicaux. Ils visionnent des vidéos, lisent les de gens qu'ils connaissent et fantasment à l'idée d'être reconnus comme de glorieux guerriers au sein de leur communauté autoréférentielle. Cette pauvreté initiale des références religieuses doit nous amener à réfléchir à une question fondamentale : quel est donc le statut de la religion dans le djihadisme ? Les observations empiriques montrent souvent que l'islam vient plus ou moins tardivement animer la conscience des acteurs, mais cela n'empêche pas de constater que, sans l'islam et, quelle que soit la pauvreté de son contenu chez les acteurs, il n'y a pas passage à l'acte ; l'action ne trouve aucun sens. Ce phénomène est puissant. En effet, on compte, selon les statistiques disponibles, environ 5 000 jeunes Européens partis en Syrie et de nombreuses tentatives de départ vers ce pays, surtout la Turquie, ont pu être neutralisées après la promulgation de lois dans de nombreux pays européens pour empêcher ces départs. Les radicalisés en France et en Europe qui ont réussi à rejoindre le théâtre syro-irakien sont devenus des combattants djihadistes. Les revers successifs de Daech posent aujourd'hui la question de leur retour. Notre collègue

étayant son propos de l'exemple d'un ex-responsable d'une cellule de déradicalisation condamné à quatre mois de prison avec sursis pour détournement de fonds, blanchiment et travail dissimulé. d'Esther Benbassa loue l'approche transversale et individualisée mise en oeuvre par les autorités au Danemark ou à Vilvoorde, en Belgique. Cette approche privilégie l'accompagnement des personnes sur leur lieu de vie, plutôt que leur déracinement au sein d'une structure, avec, notamment, une collaboration très étroite et quotidienne des services publics. Les pays européens convergent aujourd'hui sur l'idée de mettre en place un processus plus complexe que celui qui a longtemps prévalu en France, avec un traitement « au cas par cas », à la fois dans la réponse judiciaire et dans l'accompagnement en vue de la réinsertion, en ayant recours, par exemple, à des psychologues ou encore à des travailleurs sociaux. Ce modèle est celui qui est promu en Allemagne, pays qui, fort de son expérience avec les groupes d'extrême droite radicale, a très vite compris l'intérêt de l'individualisation des suivis. Alors que Daech subit une perte quasi totale de terrain en Irak et en Syrie, l'ombre du retour des djihadistes et de leurs accompagnateurs s'étend chaque jour un peu plus sur notre pays. hommes et 300 femmes, se trouvent encore en zone syro-irakienne et pourraient revenir en France ; il faut y ajouter environ 500 mineurs. La question d'un retour éventuel dans l'Hexagone, avec les risques importants que cela comporte, est donc plus que jamais d'actualité. En effet, 1 700 Français sont partis rejoindre les zones djihadistes depuis 2014. Sur ce total, 278 sont morts, mais ce chiffre est probablement sous-évalué ; 302 sont revenus en France, dont 66 femmes et 58 mineurs.

Concernant la délicate question des enfants de ces djihadistes, le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a indiqué que la plupart d'entre eux ont moins de 12 ans et que ses services étudient, avec ceux du ministère de la justice, les moyens de leur redonner un autre horizon. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a rappelé sans ambiguïté récemment : le fait, pour un ressortissant français, de se trouver dans une zone de combat est pénalement répréhensible. De plus, il est parfaitement clair que l'État français n'organisera pas le retour de ceux qui ont fait le choix de combattre la coalition. Tous les combattants qui reviennent sur le territoire national sont immédiatement soumis à une procédure pénale. C'est le cas des neuf personnes qui sont revenues depuis le début de l'année 2017. Quelles réponses donner face au retour des djihadistes français ? C'est la question que nous avons choisi de traiter ce soir. Le principe est celui d'un traitement judiciaire systématique, en retenant une qualification de nature criminelle. Il a été adopté par le procureur de la République de Paris pour tous les individus de retour d'une zone de combat. La prise en charge judiciaire des « revenants » se fait donc, depuis 2015, par un placement en garde à vue des femmes et des hommes majeurs et des mineurs combattants. Le parquet de Paris avait anticipé le phénomène des retours en durcissant sa politique pénale : jusque-là considéré comme un délit passible de dix ans de prison, le fait d'avoir rejoint les rangs de Daech est désormais un crime passible de vingt ans à trente ans de réclusion. L'objectif est clair : tous ceux qui reviennent des zones de combat doivent passer entre les mains de la justice. Après leur placement en garde à vue, le juge des libertés et de la détention peut décider d'une incarcération. Je le rappelle, à ce jour, sur les 178 hommes revenus, 120 sont en prison, ainsi que 14 femmes sur les 66 revenues. À ce propos, il faut noter que les femmes « revenantes » ont longtemps bénéficié d'un « biais de genre », au motif qu'elles auraient été embrigadées par des recruteurs masculins, mais les enquêteurs ont fini par comprendre que leur degré de radicalisation n'avait souvent rien à envier à celui des hommes. Elles sont désormais mises en examen et de plus en plus fréquemment placées en détention. Les autres, ceux qui ne sont pas incarcérés, font tous l'objet soit d'un suivi administratif des services de renseignement, soit d'un suivi judiciaire lorsque les juges ont décidé d'un placement sous contrôle judiciaire, soit d'une mesure de suivi du type du sursis avec mise à l'épreuve. Le ministère de la justice a également mis en place un dispositif d'accompagnement de ce type de personnes, afin d'assurer un suivi judiciaire renforcé de ces individus et de leur permettre de bénéficier d'un suivi individualisé. Les mineurs non combattants font eux aussi l'objet d'un suivi systématique par un juge des enfants au titre de la protection de l'enfance et sont placés dans des structures d'accueil de l'aide sociale à l'enfance des conseils départementaux. Tel est, mes chers collègues, l'état des lieux qui peut être dressé. Notre débat de ce soir

et, d'autre part, d'un suivi très individualisé. La judiciarisation est désormais systématique pour les majeurs revenant de la zone irako-syrienne, et ce dès leur arrivée sur le territoire national. la politique pénale menée à l'égard des adultes qui reviennent des terrains de combat prévoit désormais une telle judiciarisation systématique dès lors qu'ont été recueillis suffisamment d'éléments permettant d'établir que ces individus se sont rendus sur zone pour rejoindre un groupe islamiste combattant. En pratique, cela signifie que, dès leur arrivée sur le territoire français, tous les majeurs « revenants »- hommes ou femmes -font l'objet d'une mesure de garde à vue, suivie d'une mise en examen du chef d'association d'association de malfaiteurs terroristes. Ils font par ailleurs l'objet, dans la grande majorité des cas, d'un placement en détention provisoire ou, plus rarement, de mesures de contrôle judiciaire. La situation que je vous décris là est le fruit d'une évolution. En effet, jusqu'à la fin de l'année 2015, le parquet requérait la mise en examen et le renvoi de ces individus du chef d'association de malfaiteurs terroristes délictuelle. Ceux-ci avaient alors d'association de malfaiteurs terroristes délictuelle. Ceux-ci avaient alors vocation, à l'issue de l'information judiciaire, à être jugés par la seizième chambre du tribunal correctionnel de Paris, devant laquelle ils encouraient une peine d'emprisonnement de dix années.

avec l'activité réelle des organisations terroristes dont la commission quotidienne de crimes d'atteinte aux personnes sur zone ne fait plus aucun doute. Il est donc désormais requis par le parquet de Paris la mise en examen des « revenants » adultes du chef

sont tournées vers la démonstration que l'intéressé a effectivement participé sur zone, quel qu'ait été son rôle, au fonctionnement d'une organisation terroriste qui s'est livrée à des exactions ou à des actes de nature criminelle au préjudice de la population locale. À ce jour, 244 majeurs sont recensés par les services de renseignement comme étant rentrés sur le territoire national après avoir séjourné en zone irako-syrienne,

Une première catégorie regroupe un peu moins d'une quarantaine d'individus qui, après avoir fait l'objet d'une enquête judiciaire, n'ont pas été poursuivis faute, pour les enquêteurs, d'avoir réuni suffisamment d'indices de commission d'une infraction terroriste,

à être suivies par les services de renseignement afin de prévenir toute éventuelle menace. Il s'agit le plus souvent de femmes ayant séjourné peu de temps sur zone, et généralement au début du phénomène des filières irako-syriennes.

dans le cadre de procédures judiciaires. Bien entendu, toutes ces personnes, hommes ou femmes, suivies par les services administratifs ont vocation à être « judiciarisées » à tout moment, dans l'hypothèse où elles apparaîtraient comme représentant une menace.

La montée en puissance du renseignement pénitentiaire depuis sa création récente s'est accompagnée d'un renforcement de ses effectifs. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de créer trente-cinq emplois supplémentaires pour le renseignement pénitentiaire,

Depuis le début de l'année, tous les détenus radicalisés quittant la détention, que ce soit à l'issue d'une peine ou d'une mesure de détention provisoire, font systématiquement l'objet d'une « note de signalement

pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, si les individus sortants font l'objet d'une peine en milieu ouvert. Par ailleurs, les détenus sortant à l'issue d'une peine font l'objet d'un suivi judiciaire spécifique par deux juges d'application des peines spécialisés

Cette question cruciale prend de l'ampleur depuis novembre dernier et la prise de Raqqa. Nous savions qu'environ 1 700 Français avaient rejoint les zones djihadistes irako-syriennes depuis 2014. Même si Daech est en passe d'être définitivement vaincu militairement dans le secteur, ses membres terroristes demeureront actifs. Ils menacent de se diluer dans la population pour exporter le conflit, notamment en France, où les terroristes ont toujours l'oreille attentive de certains Nous savons que des Français ont pris part à des massacres et pratiqué la torture de masse. Entraînés et formés, ces individus aguerris sont des vraies bombes à retardement. Parmi les personnes déjà rentrées, 398 sont actuellement mises en examen, dont 260 placées en détention provisoire. Or, 690 djihadistes français se trouveraient encore aujourd'hui en Irak et en Syrie, avec 295 femmes et 400 enfants. Combien sont morts ? Difficile à dire ! Quelques dizaines d'adultes combattants ou leurs épouses, accompagnées de leurs enfants, seraient désormais assignés à résidence ou en prison là-bas. D'autres survivent dans la clandestinité. Leurs familles, inquiètes de les voir condamnés à la peine de mort en Irak ou en Syrie, Le 13 novembre 2017, le Président de la République a appelé à une gestion de ces retours au cas par cas. Les enfants, cet héritage empoisonné que Daech lègue à la France, ne peuvent être traités de la même manière que des criminels de guerre.

à la mise en place d'une commission d'enquête au Sénat sur la prise en charge des djihadistes français et de leur famille, en raison de procédures en cours concernant des

plus grands défis de sécurité auquel nous serons confrontés dans les années à venir. L'enjeu principal est d'identifier ces djihadistes sur le terrain dans la zone irako-syrienne. Il importe de savoir qui ils sont et ce qu'ils font, pour déterminer quand ils rentreront. Cette question du retour ne concerne pas exclusivement les djihadistes ayant la nationalité française ou une double nationalité, mais touche tous les combattants de Daech qui veulent entrer en France, quelle que soit leur nationalité. Or, pour entrer légalement sur le territoire national, il n'existe pas cent possibilités. Cette immigration est liée soit au travail, soit au regroupement familial, soit au droit d'asile. Les entrants relevant de cette dernière catégorie doivent nous intéresser particulièrement. Attention : il ne s'agit surtout pas de faire le moindre amalgame entre demandeurs d'asile et terroristes. Il serait dramatique que la menace de ces barbares nous fasse renoncer à notre vocation d'accueil et de protection des personnes victimes

Nous avons consacré notre dixième proposition à cette problématique. Aujourd'hui, la réalité nous rappelle que, une fois de plus, nous n'avons sans doute pas su anticiper de façon globale un risque annoncé. Elles sont nombreuses ces femmes jeunes, parties en quête du mari idéal et d'une vie romanesque, qui ont finalement été traitées comme des ventres à produire des enfants-soldats. Combien sont-elles à être revenues ? Combien sont-elles à vouloir rentrer ?

afin que ceux-ci retrouvent de solides repères, et préparer une réinsertion sociale ? Enfin, quelle prise en charge avez-vous prévue, madame la garde des sceaux, pour les enfants-soldats, ceux qui ont été embrigadés avant de rentrer en France ? La

La question reste ouverte.

Les situations sont diverses : mineurs radicalisés partis seuls, enfants mineurs de djihadistes embrigadés par Daech comme combattants en tant que « lionceaux du califat », ou encore, cas le plus fréquent, mineurs nés sur place ou très jeunes. Nous savons que bon nombre d'entre eux reviendront d'ici peu sur le territoire français, dont certains sont en passe de devenir de véritables « bombes à retardement Les mineurs emmenés ou nés en zones de combat ne sont pas responsables des choix de leurs parents, ni des éventuelles ignominies commises par ces barbares.

Ma question porte sur les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour prévenir toute dégradation de la situation de ces mineurs, les désengager de la violence extrémiste et favoriser leur insertion dans la société.

Quels sont les résultats de cette expérimentation ? Est-elle transposable aux mineurs ? Sinon, envisagez-vous d'autres programmes pour ces derniers ? La parole

ou l'Europe. Madame la ministre, au-delà du travail remarquable accompli par les services de renseignement, nos forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, sont-elles en mesure de découvrir et de faire remonter des éléments relatifs à ces combattants, dont on méconnaît les intentions à l'heure de leur possible retour sur notre territoire ? de leur possible retour sur notre territoire ? Par ailleurs, selon un rapport d'un organisme européen travaillant sur la prévention de la radicalisation, environ 460 mineurs français vivaient dernièrement sur le territoire contrôlé par l'État islamique, d'entre eux étant nés sur place. Leur retour pose beaucoup de questions, compte tenu des événements traumatisants, des combats ou des atrocités auxquels ils ont assisté, mais aussi du fait de leur possible enrôlement par Daech. de ces mineurs, qui ont majoritairement moins de 15 ans, tenteront de rentrer prochainement en France et pourront se noyer dans le flux des mineurs non accompagnés. De plus, à la différence des djihadistes adultes, les mineurs ne figurent pas sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Madame la ministre, comment assurerons-nous le repérage de ces enfants, et quels types de mesures de placement ou d'accompagnement psychologique appropriées seront mises en place à leur retour ? Enfin, disposons-nous, au sein des différentes structures d'accueil, de personnels et d'éducateurs formés à ces situations

pour faire un bilan sur l'ensemble des personnes qui peuvent être signalées par la DGSI, la DGSE, les services de la protection judiciaire de la jeunesse ou les procureurs,

à se radicaliser au point de commettre de tels actes sur le territoire, pour certains, ou de se rendre sur les théâtres d'opérations, pour d'autres, notamment en Syrie ou en Irak. Lors du conseil Justice et affaires intérieures de juin 2013, votre prédécesseur Mme votre prédécesseur Mme Taubira, ministre de la justice, Manuel Valls, ministre de l'intérieur à l'époque, et nos partenaires européens avaient demandé au coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, de recenser les mesures qui pourraient être prises. Depuis 2015, sur la base des propositions faites par la France, des mesures et des politiques visant à contrôler le retour de djihadistes en Europe ont été mises en place. On peut notamment citer l'instauration de contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Europe, la mise en place d'un système européen de données des passagers de vols aériens, la lutte contre la fraude aux documents d'identité, la création d'un réseau de sensibilisation à la radicalisation ou la lutte contre la propagande et l'apologie du terrorisme sur internet. Si elles vont dans le bon sens, ces mesures ne sont pas suffisantes. Des failles existent et certains dispositifs, comme le PNR, pu montrer leurs limites. L'approche européenne de la question du retour des djihadistes mérite incontestablement d'être renforcée. La France et l'Union européenne se trouvent aujourd'hui confrontées à un vrai défi. Le rapport réalisé par le réseau de sensibilisation à la radicalisation, le RAN, dénombre plus de 3 000 personnes ayant

de renforcer l'approche européenne en matière de lutte contre le retour des djihadistes. Vous avez cité à juste titre le RAN, qui joue un rôle essentiel de ce point de vue.

L'Union européenne a également adopté, le 15 mars 2017, une nouvelle directive relative à la lutte contre le terrorisme, qui vise à incriminer de manière uniforme sur le territoire européen le fait de partir à l'étranger pour y recevoir un entraînement à des fins terroristes ou de financer et organiser de tels voyages. Cette harmonisation européenne est extrêmement intéressante. Elle permettra

pour les « revenants ». Notre propre législation est déjà conforme à cette directive, qui entrera en vigueur au mois de septembre prochain. J'ai eu très récemment l'occasion de parler avec le commissaire européen chargé de ces dossiers.

les Français convertis à l'islam radical et partis faire le djihad en Irak ou en Syrie sont des djihadistes. Depuis la chute des bastions de Daech, le retour des djihadistes français est « la » question

« revenants » toute capacité de nuire à l'avenir. Nous sommes dans un État de droit et ils sont justiciables devant le droit français en fonction des preuves présentées. Or, nous disposons d'un ample arsenal juridique. Le livre IV du code pénal est dans une large mesure consacré à la criminalité organisée et au terrorisme. Le retrait de la nationalité française est prévu, en particulier à l'article 23-8 du code civil,

je suis convaincue que la répression est une arme. Mais nous sommes dans un État de droit, et tout individu qui a purgé sa peine l'a purgée

Leroy, pour la réplique. Les déçus du djihad sont, au minimum, suspects d'intelligence avec l'ennemi ou de participation à une armée étrangère. Ce sont donc des traîtres à la Nation. Le niveau de dangerosité de ces ennemis de la France est tel que l'on doit envisager des mesures drastiques pouvant aller jusqu'à la déchéance de nationalité. Il faut conclure ! Cette mesure n'a jamais été plus en adéquation avec la menace qui pèse sur nos concitoyens, aujourd'hui et, surtout, demain, après que cette peine

irako-syrienne. Dans les rangs de Daech, les combattants dits « étrangers » venus principalement de France, de Belgique, du Maghreb, mais également de Tchétchénie, sont les plus déterminés et, disons-le, les plus sadiques. sadiques. Le retour en France des familles françaises de Daech nous inquiète donc tout particulièrement et interroge notre capacité, dans un État de droit, à les prendre réellement en charge tout en les empêchant définitivement de nuire. Telle est la véritable question. C'est pourquoi nous devons travailler rapidement sur ce sujet, en toute transparence et sans tabou. Le 15 octobre dernier, sur Europe 1, Florence Parly, sans langue de bois, a donné la position des autorités : « Si des djihadistes périssent dans ces combats, »- sous-entendu, à Raqqa -« je dirais que c'est tant mieux. » Mais que fait-on de tous les autres, notamment des mineurs qui, de retour en France, sont rendus à leur famille, au sein de laquelle on cultive souvent la haine de la France, des juifs et des mécréants ? Madame la ministre, nous allons tous vous poser à peu près la même question et vous nous ferez sensiblement la même réponse ... Bâti sur un socle de principes humanistes et libéraux, l'État de droit restera-t-il impuissant face au défi de taille qui nous est aujourd'hui lancé et qui menace jusqu'à notre existence même ?

assez serrées. La plupart des hommes et des femmes qui reviennent en France sont soit placés en détention, soit soumis à un contrôle judiciaire.

cela devient extrêmement improbable aujourd'hui, vu l'extrême vigilance de l'ensemble des services de renseignement. Je n'ai pas à livrer les secrets des conseils de défense, mais je puis vous assurer que, chaque semaine,

dans notre État de droit- j'insiste sur ce terme -, ne faudrait-il pas mettre en place une nouvelle stratégie et de nouveaux outils en termes de détection et de déradicalisation ?

à des actions terroristes. En outre, la question se pose de savoir si ces personnes ont agi librement ou sous contrainte. Il est nécessaire de disposer d'informations fiables et de preuves à cet égard. Pouvez-vous, madame la garde des sceaux, nous préciser quels moyens sont mis en oeuvre à cet effet par votre ministère et par les juridictions compétentes ? Par ailleurs, un certain nombre de personnes de retour de Syrie ou d'Irak se présentent comme des repentis et affirment n'avoir pas mesuré au départ la nature terroriste des agissements qu'ils ont découverts sur place. D'autres déclarent avoir été radicalisés et avoir adhéré à cette radicalisation, mais en être revenus, et choisissent de la dénoncer. Certains centres actions de sensibilisation et des formations contre la radicalisation ont pu faire appel à de tels repentis pour éclairer des jeunes ou moins jeunes tentés par ces aventures à caractère terroriste et les dissuader

comme une intention immuable ? Que peut-on espérer du travail des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des pédopsychiatres ? Aucun processus ne semble aujourd'hui porter le moindre fruit. Cet état de choses impose pour le moins une grande vigilance. Je vous serais reconnaissant, madame la garde des sceaux, de bien vouloir nous informer de l'analyse de votre ministère à cet égard et de la manière dont ce dernier, et toutes les instances compétentes, appréhendent ce phénomène des repentis. La parole

plupart des ressortissants français, mineurs comme majeurs, qui ont été capturés sur zone en Syrie sont remis par les factions armées aux autorités turques, voire aux autorités irakiennes. Lorsqu'ils sont appréhendés par les autorités turques après franchissement de la frontière, les ressortissants français sont pris en compte, sur un plan administratif, en vertu du protocole franco-turc

Plus de 300 personnes sont déjà revenues des zones djihadistes, dont 66 femmes et 56 mineurs, âgés pour la plupart de moins de 12 ans. Les services de renseignement estiment à plus de 400 le nombre de mineurs français qui seraient encore sur place. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a permis, sous l'impulsion du Parlement, de « judiciariser » le retour des femmes. Aujourd'hui, elles sont placées en détention provisoire, le temps que leur dossier soit instruit. Pendant ce temps, les enfants sont confiés aux services départementaux d'aide sociale à l'enfance, comme des orphelins classiques, avant que le juge des enfants ne se prononce sur un type de placement soit en foyer, soit en famille d'accueil, soit chez un proche. Or, comme le souligne le procureur de la République, ces enfants peuvent devenir de « véritables bombes à retardement ». L'enjeu de leur prise en charge est donc double : reconstruire ces enfants traumatisés et assurer la sécurité des Français. Toutefois, chacune des trois possibilités de placement que j'ai citées comporte des écueils. Dans les foyers,

À l'heure où l'État islamique recule, la question du retour des femmes et de leurs enfants devient de plus en plus préoccupante. Son traitement demande des moyens et une attention particulière au vu de sa spécificité. Début septembre, le Président de la République avait annoncé son intention de revoir la prise en charge de ces enfants, à partir de propositions formulées par les ministères de la justice, de la santé et de l'intérieur, « d'ici à la fin de l'année ». Madame la garde des sceaux, où en sont les travaux sur ce point ? Quelles sont les premières pistes d'action envisagées ?

âgés de moins de 10 ans. Lorsqu'ils arrivent en France, ces mineurs font systématiquement l'objet d'une ordonnance de placement provisoire puis d'une saisine d'un juge des enfants, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.

Le juge des enfants sollicite une évaluation très précise de leur situation par les services de la protection judiciaire de la jeunesse pendant six mois. Par la suite, le mineur va faire l'objet d'une prise en charge et d'un accompagnement renforcés, qui associent les compétences des services de la PJJ et celles des conseils départementaux. Lorsqu'ils sont placés, ils font l'objet, et c'est nouveau, d'une double mesure

La menace est élevée, elle ne faiblit pas malgré la mise en oeuvre d'un arsenal législatif profondément renforcé ces dernières années. Aujourd'hui, nous devons faire face à un réel problème, celui des retours de djihadistes français sur notre sol. L'État estime à plus de 100 le le nombre de ressortissants français encore présents dans les territoires irakien et syrien. On compte également près de 300 femmes et une trentaine de mineurs de plus de 15 ans. Madame la garde des sceaux, ceux qui ont quitté notre pays ont décidé de prendre les armes contre leur propre peuple. Ils ont fait le choix de la mort et de la barbarie. Ils doivent être jugés dans les pays qui les détiennent. Pourquoi la France devrait-elle prendre le risque de rapatrier ces individus et de rouvrir des plaies encore profondes et douloureuses ? La vie est une succession de choix qu'il convient d'assumer les leurs sont sûrement les pires qui existent, mais cela ne les exonère pas de les assumer pleinement. Reste la question des enfants : ils ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables ou complices des actes de leurs parents. La France doit, au cas par cas, organiser leur retour. C'est son honneur que de le faire. N'oublions pas non plus la question sensible du retour des mères de famille.

Ne soyons pas naïfs ; nous ne pouvons pas présumer que, parce qu'elles sont femmes et mères, elles ne sont pas profondément imprégnées de l'idéologie djihadiste. Elles sont souvent le moteur idéologique dans le couple, l'homme étant davantage attiré par la dimension combattante.

en les mettant hors d'état de nuire ? Il faut conclure ! Qui porterait la responsabilité de leur influence idéologique au sein de nos prisons, qui sont déjà des nids de radicalisation ?

Vous opposez l'État de droit, que nous défendons tous et qui par essence est un État rationnel, fondé sur le respect de la règle, à des

Ainsi, de nombreuses interrogations pèsent sur l'efficacité et la fiabilité des résultats de certaines institutions, comme l'ont montré les polémiques de cet été sur le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam de Mme Dounia Bouzar. Ces échecs tiennent à la logique même qui sous-tend

D'autres pays l'ont bien compris : des expériences réussies en Norvège, aux Pays-Bas ou en Allemagne pourraient nous inspirer. Ces pays fondent leur action sur la volonté politique d'intégrer les communautés musulmanes locales et des acteurs sociaux variés, sans stigmatisation ni mise au ban de la société. Leur approche est englobante ; elle prend en compte l'environnement familial, social, scolaire, culturel et géographique, pour se rapprocher d'un traitement au cas par cas. Ce type d'approche devrait faire l'objet d'une harmonisation à l'échelle européenne, sur la base d'un partage des meilleures pratiques. Les résultats du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation, le RAN, sont insuffisants, comme les moyens alloués à cette politique dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure. Or, face à la menace transnationale que constituent le retour des djihadistes européens et les phénomènes de radicalisation, l'Union européenne doit jouer collectif et être en première ligne. Ma question, madame la garde des sceaux, est la suivante

La République En Marche. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur du débat disposera

que notre assemblée débatte ce soir de la COP23 et, plus généralement, de l'état des engagements et des initiatives pris par notre pays en matière de lutte contre le changement climatique ? Tout simplement parce que la lutte contre le réchauffement climatique est le combat majeur de notre temps, comme l'a si justement rappelé le Président de la République,

mal, si mal que, le 13 novembre dernier, plus de 15 000 scientifiques, issus de 184 pays, ont averti l'humanité entière par ces mots : « Bientôt, il sera trop tard. » Notre planète va mal, et même de plus en plus mal. C'est une évidence qui doit être répétée, même si certains, et non des moindres, s'évertuent encore à la nier. Le constat des climatologues est alarmant ; les faits concordent dramatiquement, au point que les relevés les plus récents sur l'évolution du climat mondial soulignent que nous nous inscrivons actuellement dans le pire des scénarios pourtant actualisés il y a moins de trois ans. Il ne passe pas un jour sans qu'une nouvelle information ne vienne témoigner, très concrètement, de l'impact du réchauffement climatique sur nos écosystèmes fragiles et sur la vie des hommes sous toutes les latitudes de notre planète. Déclin rapide de la riziculture dans le delta du Mékong en raison de la remontée des eaux salines de la mer dans les terres cultivées, détachement soudain d'immenses surfaces de glace de mer en Antarctique, zone pourtant longtemps considérée comme la plus préservée du réchauffement climatique

avait débouché sur un accord international, qualifié d'historique, par lequel 197 États s'étaient engagés à limiter la hausse des températures mondiales à 2°C, voire à 1,5°C, à l'horizon de la fin du siècle.

déjà, le président Chirac prononçait ces fameuses paroles : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Treize ans plus tard, Barack Obama entamait la présentation de son plan pour l'environnement par cette phrase : « Nous n'avons qu'une planète : il n'y a pas de plan B. Hier, dans le cadre du, le Président Emmanuel Macron dressait un constat encore plus inquiétant : « Nous sommes en train de perdre la bataille. » Le but premier de ce sommet, organisé par la présidence française, était précisément de dépasser le temps du constat et des engagements diplomatiques formels,

fort opportunément le système des conférences sur le climat ; il ne le concurrence pas. La COP23, qui s'est achevée le 17 novembre dernier à Bonn, et la future COP24 de Katowice, en Pologne, ne peuvent produire que des accords multilatéraux s'inscrivant dans une démarche onusienne, soumise tant aux contraintes des négociations diplomatiques qu'au bon vouloir des dirigeants des pays signataires. Certes, au sortir de la COP23, quelques avancées positives sont à noter. Nous ne pouvons qu'accueillir avec bienveillance la mise en place d'une plateforme sur les savoirs et les connaissances des peuples autochtones une aide dans la lutte contre le bouleversement du climat. Cette mesure s'adresse à 300 millions d'individus qui voient leurs terres et leurs vies directement menacées par le changement climatique. Nous nous félicitons également de la création d'un groupe de travail sur la sécurité alimentaire, en vue de repenser des systèmes industriels dévastateurs et de renforcer les mesures visant à protéger l'agriculture paysanne. Il en va de même de la mise en place du plan d'action pour l'égalité des sexes et du lancement d'une alliance pour la sortie du charbon par le Royaume-Uni et le Canada,

Les pays les plus vulnérables sont partis de cette conférence sans nouvelle annonce de financements pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Si ces conférences sont nécessaires, force est de constater que les objectifs seront atteints bien trop lentement. la spécificité de la COP23 était de progresser sur la définition de règles d'application de l'accord de Paris de 2015, mais ces dernières ne pourront être finalisées que l'an prochain. Ainsi, de 2015 à 2018, trois années se seront écoulées avant qu'une quelconque mise en oeuvre de l'accord de Paris soit effective.

regroupe 86 agglomérations représentant plus de 600 millions d'habitants, 25 % du PIB mondial et 70 % des émissions de gaz à effet de serre.

pour lutter contre le réchauffement climatique. Los Angeles, qui doit faire face à des incendies monstrueux dus à la sécheresse, a bien conscience que le changement climatique est désormais une réalité quotidienne. Concernant le secteur privé, je veux rappeler ici que l'engagement pris par de grandes entreprises ou institutions financières en matière de lutte contre le réchauffement climatique est capital. Il sera, à l'avenir, absolument déterminant pour atteindre les objectifs fixés à Paris il y a deux ans.

ou tout imposer par une forme de coercition réglementaire. Le combat contre le changement climatique n'est pas que de nature politique ; il s'agit bien d'un combat culturel et civilisationnel, qui doit mobiliser tous les acteurs de la société, ceux qui, par intérêt immédiat, y sont modérément sensibles, si nous voulons nous donner une chance de le remporter. Quoi qu'on en dise, le monde des grands acteurs de l'économie et de la finance est en train d'évoluer très sérieusement en matière de responsabilité climatique et environnementale. La preuve la plus éclatante de ce changement tient croissante prise, ces trois dernières années, par le mouvement de désinvestissement dans le domaine des énergies fossiles dans lequel se sont engagés certains groupes financiers et de grandes institutions publiques, parapubliques ou privées. Lancé en 2007 par l'écrivain et journaliste américain Bill McKibben, le mouvement 350.org, qui incite précisément au désinvestissement désinvestissement financier des entreprises des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre, rencontre un succès inattendu. Les investisseurs sont désormais de plus en plus attentifs

aujourd'hui, dans l'action, dans la transformation de nos modes de vie et de nos comportements, mais aussi de notre économie, de nos façons de travailler et même de penser.

L'énergie nucléaire reste absolument essentielle, notamment pour assurer la sécurité d'approvisionnement pour tous les Français, Français, mais nous voulons peu à peu réduire sa part, ou en tout cas rééquilibrer notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Les transports sont

et les petites îles, qui représentent environ 40 % des projets et 30 % des engagements financiers, n'ont pas été pénalisés en termes de volume d'engagements. Un processus d'approbation simplifié pour les petits projets non risqués sur les plans environnemental et social a été validé par le conseil au mois d'octobre 2017.

terme des mandats des membres du conseil, à la fin de 2018, devra être l'occasion de repenser le mode de gouvernance du fonds. Nous nous y attacherons en soutenant le renforcement du secrétariat

pour évoquer le financement de la transition énergétique. Encourageant, car cette rencontre, même si on ne comprend pas bien pourquoi elle ne pouvait pas se tenir dans le cadre de la COP23, le mois dernier, n'a guère de précédent. Curieux, car il est difficile de concevoir que la grande finance, principale responsable du dérèglement climatique, puisse contribuer sans règle à sa résorption. En effet, si la planète est aujourd'hui à ce point en péril, c'est la conséquence directe de la recherche permanente de la rentabilité, de l'hyperfinanciarisation de notre économie et de la marchandisation du vivant. Madame la secrétaire d'État, si nous savons bien qu'aucun espoir ne sera permis sans une mobilisation de toutes et tous, en particulier des acteurs économiques, vous comprendrez aisément les réserves que nous inspire cette finance dite « verte Nos doutes ont été confortés par le rapport rendu public par l'association ATTAC, confirmant que ces obligations vertes, les, relèvent trop souvent de l'escroquerie. En effet, aujourd'hui, rien ne garantit que ces investissements soient climato-compatibles. Ces obligations ne sont ni contrôlées ni régulées. Il en est ainsi des obligations émises par Repsol, multinationale du pétrole, qui visent en réalité à prolonger la durée de vie des raffineries

Seulement 25 % de ces obligations sont aujourd'hui certifiées, c'est-à-dire répondent directement à leur objectif premier de préservation de l'environnement. C'est peu. Madame la secrétaire d'État, quelles mesures pensez-vous pouvoir prendre pour nous garantir que, demain,

Nous avons vu des pays moins mobilisés, plus attentistes, moins motivés pour s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, on a aussi remarqué la présence d'acteurs américains, notamment des maires de grandes villes, des responsables d'universités, de centres de recherche, d'entreprises, d'associations

des conséquences du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Quelques heures après la décision du président Trump, le Président de la République s'est adressé, en anglais et en français, à la planète entière.:

que l'Afrique ne contribue que dans une mesure infime aux émissions de gaz à effet de serre, avec moins de 4 % des émissions totales, et que « le financement d'un plan stratégique de développement en Afrique est une question de réparation des dommages historiques et d'équité à même de conjurer les effets négatifs des déséquilibres climatiques sur le continent cet appel unanime s'interrogeaient par ailleurs sur la tenue des engagements financiers à l'égard du Fonds vert pour le climat. Cet instrument financier devait promouvoir l'énergie verte dans les pays les moins avancés ; le retrait des États-Unis est une source d'inquiétude. à attendre les 100 milliards de dollars par an promis à partir de 2020, le cauchemar climatique, lui, n'attend pas : montée des eaux aux îles Fidji, disparition de terres, sécheresses dans l'histoire de la Corne de l'Afrique, ouragans ne laissant plus un arbre debout aux Îles Vierges ... C'est là toute l'injustice de la situation : les moins responsables sont les plus vulnérables et les plus touchés. Les parlementaires de ces pays en voie de développement attendent des actions et se disent las

N'oublions pas qu'aujourd'hui 300 millions de personnes, notamment les habitants des petits États insulaires- les îles Maldives, Marshall, Fidji ... -, voient leur quotidien, leur histoire, leur vie même directement menacés par ce bouleversement climatique. Oui, des États vont purement et simplement À Bonn, des milliers de manifestants ont défilé pour la lutte contre le changement climatique. Il s'agissait d'accentuer la pression sur les dirigeants que nous sommes. J'ai moi-même été frappée et émue par l'appel des parlementaires africains, qui ne demandent pas l'aumône, mais attendent un investissement à la hauteur de nos responsabilités.

la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, la France a pris hier des engagements importants en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement et les pays les moins avancés.

Dans ce combat, le monde des entreprises a des responsabilités ; il a aussi des engagements. Voilà quelques jours, huit grandes entreprises françaises ont décidé d'investir 50 millions d'euros pour lutter contre le changement climatique. Hier, entreprises françaises, représentant 6 millions d'emplois dans le monde, ont annoncé leur ambition de réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises engagées dans cette démarche proposent d'investir dans les secteurs des énergies renouvelables,

doit être un levier providentiel pour gérer la transition vers une économie décarbonée. En effet, il suffirait d'accroître la capacité naturelle des sols à stocker le carbone de seulement 4 pour 1000 annuellement pour compenser une part importante des émissions mondiales de CO2.

peu à peu, mais le plus rapidement possible -, de changer de paradigme. L'initiative « 4 pour 1000 », lancée lors de la COP21 par la France, est véritablement emblématique de ce que nous devons promouvoir pour accélérer la transition écologique dans le secteur de l'agriculture. Le but de cette initiative est d'accroître la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Les trois principaux objectifs sont d'assurer la sécurité alimentaire en accroissant la fertilité des sols, d'adapter l'agriculture au changement climatique, mais aussi, bien sûr, de contribuer à l'atténuation du changement climatique, notamment grâce aux services rendus aux écosystèmes, comme vous le soulignez dans votre question, monsieur le sénateur.

Cette feuille de route prévoit l'élaboration d'un référentiel d'évaluation des projets et des actions, un programme de recherche, une plateforme collaborative, ainsi qu'un centre de ressources.

terres. Une réunion de grande ampleur du Forum et du Consortium a été organisée en partenariat avec l'Allemagne, à Bonn, lors de la COP23. Comme

affirmé hier que nous devrons être capables, collectivement, d'être aussi ambitieux pour sauver le climat que nous l'avons été pour sauver les banques en 2008. Nous avions alors mis 1 000 milliards d'euros Il faut savoir être à la hauteur de ses ambitions. Nous partageons totalement ce point de vue. La

ont finalement été les négociations visant à faire appliquer l'accord de Paris sur le climat signé lors de la COP21. Pour rappel, l'indéniable succès de la COP21 est à la mue de la diplomatie écologique, qui est passée d'une démarche à une méthode fondée sur des contributions volontaires. Le travail accompli pour obtenir l'accord de Paris

Nous ignorons encore comment seront évalués les résultats et comment le fonds de 100 milliards de dollars destiné aux pays en voie de développement sera constitué. L'organisation du dialogue dit « de Talanoa » doit permettre aux États d'accroître leurs ambitions pour contenir le réchauffement climatique sous les deux degrés.

va-t-elle rehausser ses objectifs ou les stabiliser ? La diplomatie française va-t-elle privilégier un rehaussement généralisé des contributions étatiques ou se concentrer sur les moyens de contrôler les engagements actuels ? Enfin, et surtout, pensez-vous, que le seuil de l'irréversible a été franchi

Elle mobilisera également trois milliards d'euros entre 2016 et 2020 pour le développement des énergies renouvelables en Afrique. Vous le voyez, monsieur le sénateur, la France, au-delà de son engagement en faveur du verdissement de la finance, contribue également

Neutralité carbone et développement économique font bon ménage. L'engagement du monde économique est à cet égard significatif et enthousiasmant, car, en réintroduisant de la vision du sens dans les décisions de court terme, il pose de nouvelles fondations pour notre avenir économique collectif. Il crée un cadre pour l'innovation et pour des ruptures technologiques qui participeront à la construction d'un monde sans pollution. Ce cadre est non plus une contrainte, mais une émancipation. Cette émancipation impose que nous remettions au coeur du projet économique de notre pays, de l'Europe et du monde, les principes de l'économie sociale et solidaire, car l'entreprise, si elle joue un rôle majeur dans nos sociétés, parce qu'elle crée des emplois et produit de la richesse, ne peut s'extraire des travers de la mondialisation, de certains égoïsmes qui conduisent au creusement des inégalités. Il semble que le Gouvernement veuille faire évoluer l'objet social des entreprises, qui ne peut plus être le simple profit, sans considération aucune pour les femmes et les hommes qui travaillent, sans regard sur les désordres environnementaux. Cette réforme devrait vraisemblablement conduire à modifier le code civil, afin que les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire, cette économie pionnière, qui

c'est non seulement notre avenir collectif et notre capacité à développer un capitalisme raisonné et une croissance durable de nos activités, mais aussi, et surtout, l'attractivité même de nos entreprises. La

dans l'intitulé du ministère ... La transition ne pourra pas être écologique si elle n'est pas solidaire ! Si elle n'est pas solidaire, il sera plus difficile encore d'atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. C'est pour cette raison, notamment, que nous avons lancé un grand chantier en matière d'économie circulaire. Nous voulons que, à terme, l'économie circulaire devienne plus

L'économie circulaire représente aujourd'hui près de 800 000 emplois. Si nous respectons les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment celui de recycler 100 % des plastiques et de

pour la société. Tel est le projet de société que nous portons. Nous devons transformer

Cependant, l'ensemble des ONG estime qu'il est vide et qu'il s'agit d'une simple tentative de désamorcer la large opposition que suscite ce traité.

Le CETA, comme tout accord commercial, fait passer le commerce et les profits avant la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Non seulement il ignore cette urgence, mais il aggrave le phénomène. selon la Commission européenne, le CETA accroît les émissions de gaz à effet de serre, du fait notamment du développement des échanges commerciaux. Le CETA organise la libéralisation tous azimuts. Il ne prévoit aucune exception dans le secteur de l'énergie. Bien au contraire, il privilégie le commerce traditionnel des matières premières, notamment des sables bitumineux, au détriment du déploiement des énergies renouvelables, lesquelles ne sont même pas mentionnées dans l'accord. Le CETA est en totale contradiction avec l'article 2 de l'accord de Paris,

la commission Schubert, que le Président de la République et le Premier ministre ont chargée d'évaluer

entreprises, qui sont une part essentielle du tissu économique de la France.

L'affaire était pourtant bien engagée puisque la tenue de la COP21 officialisait la reconnaissance mondiale des dangers et des conséquences irrémédiables du réchauffement climatique. Mais nous le savons, les prévisions les plus pessimistes des climatologues ont d'ores et déjà été atteintes. Nous sommes à l'aube d'une crise majeure, notamment en ce qui concerne l'eau. Entre impératifs climatiques et tiraillements politiques, la COP23 est revenue sur les enjeux essentiels que sont le financement des aides aux pays en développement, les gaz à effet de serre, la pollution des eaux, ou encore les défis énergétiques. Cependant, la question pourtant centrale et fondamentale de la croissance ininterrompue de la population mondiale n'est toujours pas évoquée directement. Lundi 13 novembre 2017, plus de 15 000 scientifiques de 184 pays ont publié dans la revue une tribune intitulée « Avertissement à l'humanité ». entre autres des mesures démographiques comme la réduction du taux de fécondité et la détermination d'une taille de population humaine soutenable. En effet, la population continue d'augmenter, et le scénario moyen prévoit que nous serons près de 10 milliards en 2050, soit une augmentation de près de 30 % par rapport aux 7,5 milliards actuels. Ma question est la suivante : la COP23 a mis en lumière le travail qu'il reste à fournir pour appliquer l'accord de Paris.

Monsieur le sénateur, vous posez la question difficile et essentielle du lien entre développement économique et lutte contre le changement climatique. Le Gouvernement, comme d'ailleurs

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, malgré le cri d'alarme lancé par la communauté scientifique mondiale durant la Conférence des Parties réunie à Bonn, ce que l'on retiendra de la COP23, c'est la chaise vide du président des États-Unis. Le retrait unilatéral décidé par Donald Trump semble en effet avoir enrayé le processus lancé par la France en 2015. À l'inverse, il semble que le Président de la République soit fermement engagé à mener tous azimuts la lutte contre le réchauffement climatique. À bien des égards, le pour le climat d'hier ressemble à une séance de rattrapage de la COP21, qui, mis à part quelques engagements sur le charbon, est restée en deçà de ses promesses. quelles sont les avancées concrètes de ces cérémonies riches en déclarations d'intention ? Il semble que la Banque mondiale ait promis hier d'arrêter de financer l'exploitation

Le soutien international à une agriculture respectueuse de son environnement pourrait constituer l'une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, tout en répondant à des enjeux sociaux, économiques et alimentaires de premier plan. De l'aveu même de la Banque mondiale, les investissements dans l'agriculture sont plus efficaces que tout autre.

Que vous le trouviez satisfaisant ou non, il a le mérite de poser un cadre clair et ambitieux, compte tenu du nombre d'États qui ont signé

cinq milliards d'euros par an en 2020, dont un milliard d'euros seront consacrés directement à l'adaptation au changement climatique. L'agriculture est un axe absolument essentiel de la politique de lutte contre le changement climatique, mais aussi d'une politique

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, hier, la France a reçu de nombreux chefs d'État afin de se pencher au chevet de la planète Terre et de constater l'étendue des dégâts. Les grands pollueurs ne sont pas venus à Paris, le changement climatique étant sans doute jugé comme secondaire par leurs dirigeants ... Comme par le passé- je me souviens des déclarations de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » -, notre pays veut prendre la main sur la scène internationale et montrer l'exemple en matière de transition écologique et énergétique. En France, l'espace montagnard couvre environ un cinquième du territoire national, soit 124 000 kilomètres carrés d'espaces préservés, de réservoirs d'eau, de réserves de biodiversité, de biodiversité, que certains, surtout ceux qui n'y vivent pas, sont tentés de transformer en véritables sanctuaires. Or les montagnes françaises, et les Alpes en particulier, sont aussi des espaces de vie, où il existe une activité économique, fondée essentiellement sur le tourisme.

Les habitants de la montagne sont bien conscients du patrimoine naturel et environnemental qu'ils ont entre les mains. C'est pourquoi il est inutile de multiplier les interdictions, les restrictions et les surréglementations à la montagne.

dans chaque territoire. Notre plan Climat vise la neutralité carbone d'ici à 2050. Cela suppose de changer nos modes de production, nos modes de consommation, mais aussi

Mon collègue Sébastien Lecornu travaille au contrat de transition écologique, qui vise aussi à trouver des solutions

une peine économique, puisqu'il existe une distorsion de concurrence ; une peine écologique, puisque nous allons favoriser une production polluante et l'importer par des transports énergivores. Vous conviendrez donc que notre volonté de nous montrer exemplaires dans la lutte contre le réchauffement climatique en prend un sacré coup ! Pourtant, cet effort est nécessaire. À l'heure où les échanges et les transports de marchandises très polluants vont s'intensifier, notamment avec le traité CETA et les discussions à venir avec les pays du MERCOSUR, nous sommes en droit de nous inquiéter, surtout pour notre santé. Ainsi, à l'échelle de nos territoires et de la France, il faut que nous puissions privilégier les initiatives locales et consommer les produits qui en sont issus, pour moins polluer. Avec du chauvinisme, et pour plaisanter un peu, je vous

Cela dit, madame la secrétaire d'État, comment comptez-vous prendre en compte cette augmentation des échanges polluants dans notre lutte commune contre le réchauffement climatique ? La parole la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, contrairement aux accords passés, qui ne traitaient que des droits de douane, les accords nouvelle génération » que négocie l'Union européenne comportent des dispositions sur les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les standards et la coopération réglementaire, y compris dans le domaine environnemental.

par ailleurs la promotion dans d'autres accords commerciaux, notamment celui entre l'Union européenne et le MERCOSUR. Nous voulons par exemple promouvoir le respect effectif du principe de précaution, tel qu'il est prévu au sein des traités Nous souhaitons aussi que soit préservée la capacité des États à réguler pour des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière environnementale. Nous prônons d'ailleurs une mention explicite de l'accord de Paris. Nous encourageons ensuite les engagements à réduire les émissions du transport maritime et aérien et soutenons les initiatives multilatérales en la matière. Nous plaidons enfin en faveur de la soumission des chapitres de développement durable des accords en cours de négociation au mécanisme générique de règlement des différends de l'accord, comme c'est le cas pour tous les autres chapitres.

Voilà deux ans, le 16 novembre 2015, nous votions ici, dans cet hémicycle, à l'unanimité, une proposition de résolution visant à réaffirmer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d'un accord mondial ambitieux pour le climat. pour le climat. Avec ce texte, les sénateurs ont délivré deux messages : premièrement, les territoires sont prêts à assumer leur part d'universalité ; deuxièmement, les solutions de préservation de nos ressources naturelles existent aussi à l'échelon local. C'est toujours d'actualité. Membres du groupe socialiste et républicain du Sénat, nous avons répondu présent pour soutenir toutes les initiatives, elles aussi concrètes, visant à promouvoir la sobriété énergétique et la transformation des modes de production. Puisque nous sommes à l'heure de la concrétisation et de la responsabilisation de tous les acteurs, je crois particulièrement indispensable que nous transformions aussi les modes de déplacement quotidien et que soit menée une politique d'aménagement du territoire qui prenne en compte en permanence cette exigence universelle de lutte contre l'élévation mondiale de la température terrestre, la cohérence étant un gage d'efficacité dont nous avons besoin. À ce titre, la préservation des sites d'équipement et de service public de proximité, notamment en milieu rural, me paraît une vraie nécessité, qu'il s'agisse des établissements scolaires, des services de médecine de proximité, ou, plus largement, des services au public. Il nous faut promouvoir un effort et un engagement conjoint et cohérent.

la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, dans les territoires ruraux, compte tenu de l'offre réduite en transports en commun, la dépendance à la voiture individuelle reste très forte pour la mobilité quotidienne. Je le disais tout à l'heure, pour venir d'une circonscription rurale et avoir grandi dans une zone rurale, je sais combien nous sommes dépendants de la voiture et combien la question des transports est absolument cruciale pour notre développement économique à tous. De fait, les transports du quotidien en zone rurale émettent bien de CO2

Le développement des mobilités partagées sous diverses formes est également encouragé, car il s'agit d'une piste intéressante pour les zones rurales. Cela a fait l'objet de discussions particulièrement approfondies dans le cadre des assises de la mobilité. Il faut maintenant trouver les bons leviers pour lever les freins économiques, juridiques, mais aussi tout simplement pratiques, pour mobiliser les acteurs, les collectivités Des outils existent déjà, comme les plans de mobilité, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mais il faut passer à la vitesse supérieure. Sur le plan international également, nous avons uni nos forces en lançant une

Et parce que c'est une affaire de science, nous comptons sur le progrès technique pour relever le défi climatique. Il a beaucoup été question d'argent pendant cette COP23, avec l'alimentation du Fonds vert pour les pays en développement. Soyons conscients néanmoins que tous les pays, développés ou non, ont besoin de financements. se divise en trois sous-questions. À quand un ITER des énergies renouvelables ? À quand un ITER du stockage de l'électricité ? À quand un ITER du recyclage, notamment des métaux ? Toujours au sujet de la distinction entre pays développés et pays en développement, je ne comprends pas bien les propos du Président de la République, lorsqu'il déclare que « les pays riches ont imposé au monde leur modèle industriel ; aujourd'hui il leur est interdit d'imposer au monde leur propre tragédie ».

Même si nous le dénonçons avec force, n'oublions pas que, si les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, c'est aussi pour ne pas donner un droit à polluer à leurs concurrents commerciaux.

Or certaines associations présentes et bruyantes lors de la COP n'ont qu'une formule à la bouche : agroécologie paysanne. Quelle est votre définition de l'agroécologie paysanne ? Partagez-vous cet avis ? Enfin, vous engagez-vous à soutenir les différents autres modèles agricoles quand ils allient dans leurs pratiques technicité, productivité et développement durable ?

Elle se conçoit comme l'utilisation au maximum de la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Elle s'appuie ainsi sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes, qu'elle amplifie, tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Bien sûr, comme je le précisais, d'autres modèles sont à soutenir. Il existe déjà des outils réglementaires pour inciter changement de pratiques. Ce sont notamment les mesures agroenvironnementales et climatiques, ainsi que les aides à la conversion à l'agriculture biologique, qui relèvent de financements européens et nationaux.

Force est de constater que la France n'est pas au rendez-vous qu'elle s'était fixé. Elle est aujourd'hui largement distancée par ses voisins européens. Près de 4 000 éoliennes sont aujourd'hui installées au large des côtes européennes, et la France, qui possède plus 3 400 kilomètres de façade maritime, n'en a encore aucune en fonctionnement. Les premiers appels d'offres ont été lancés en 2011 et, en dépit d'une première simplification relative aux juridictions de recours, les projets tardent à se concrétiser dans les faits. De plus, la rigidité de la procédure impose aux industriels de figer une technologie, alors que, grâce à l'innovation, de nouveaux modèles de machines plus performantes et plus puissantes sont disponibles. Dans le domaine de l'hydrolien, qui constitue un marché de niche, la France possède un potentiel de plusieurs gigawatts. Les énergéticiens et turbiniers sont dans l'expectative. Des démonstrateurs ont été éprouvés et des fermes-pilotes sont en cours de réalisation, mais l'absence immédiate d'appels d'offres pour des fermes commerciales obère toute visibilité pour élaborer des schémas industriels permettant de rationaliser la production, donc de diminuer les coûts. lors des Assises de l'économie de la mer, le Gouvernement a affiché la volonté de revoir les procédures en organisant lui-même le débat public et en déposant des « permis enveloppes » au titre de la loi sur l'eau et de l'occupation du domaine public maritime. Ces permis enveloppes permettraient de lancer des appels d'offres purgés de tout recours et de transférer ainsi aux lauréats les différentes autorisations. Madame la secrétaire

la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou PPE, fixe un objectif de 3 000 mégawatts d'éolien posés en mer en fonctionnement et jusqu'à 6 000 mégawatts attribués à l'horizon 2023.

En amont de l'appel d'offres, l'État prendra dorénavant à sa charge l'ensemble des études préalables, par exemple les études techniques et les analyses de l'état initial, en vue de les transmettre aux candidats. Il organisera le débat public afin de déterminer la zone spécifique de l'appel d'offres. Il est également prévu, dans le projet de loi pour une société de confiance, que les autorisations nécessaires pour les énergies renouvelables en mer soient remises sous la forme d'un « permis enveloppe L'objectif de ces mesures est double : d'une part, accélérer la mise en oeuvre des projets, tout en réduisant leur coût, ce qui est un véritable enjeu ; d'autre part, à travers l'organisation du débat public par l'État

Ce nouveau cadre sera pleinement applicable aux prochains appels d'offres annoncés lors des Assises de l'économie de la mer, notamment à l'appel d'offres éolien posé à Oléron qui sera lancé en 2018.

la thématique de l'eau prend de plus en plus d'ampleur au sein des négociations internationales sur le climat. L'eau est vitale pour les hommes, ainsi que pour l'équilibre des écosystèmes, et elle est parfois un enjeu géopolitique. C'est la première ressource concernée par le dérèglement climatique, des catastrophes naturelles lui sont liées. Enfin, elle est centrale pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. L'accord de Paris, en donnant une place significative au volet « adaptation au changement climatique », a permis au secteur de l'eau de prendre un nouvel essor. Je vous rappelle que 93 % des contributions nationales qui comprennent ce volet ont identifié l'eau comme priorité. L'eau est au coeur d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux : accès à l'eau potable, assainissement, hygiène, gestion des risques, agriculture, gestion intégrée des ressources en eau. Cette volonté d'intégrer l'eau dans le programme d'action climatique prend de l'ampleur, notamment grâce à la montée en puissance de la société civile, fortement mobilisée lors de la COP22, pour la première journée d'action mondiale pour l'eau. Le problème évoqué lors de la COP23 reste le financement, qui nécessiterait d'être multiplié par trois, pour atteindre 255 milliards d'euros par an, faute de quoi serait mis en péril l'objectif du développement durable numéro 6, à savoir un accès à l'eau salubre et à l'assainissement pour tous. Aussi, je pense que l'eau doit être intégrée dans les grands secteurs, tels que l'énergie, la sécurité alimentaire ou encore la santé, et devenir la grande priorité des politiques nationales, notamment celles de la France. Au congrès des maires, le ministre d'État Nicolas Hulot a rappelé que la politique de l'eau française était un modèle « unique au monde ». Aussi, exportons-la, valorisons-la au sein des négociations internationales ! De plus, nous avons de très belles entreprises dans ce secteur : des start-up, des PME, des grands groupes. La tenue des Assises de l'eau en 2018

Monsieur le président, monsieur le sénateur, pour la première fois, une COP était présidée par un petit État insulaire, les îles Fidji,

En parallèle, l'eau joue un rôle primordial dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique avec l'hydroélectricité comme vaste mode de production propre d'électricité. La thématique de l'eau a été particulièrement visible en zone « Bonn » lors de la journée « eau » de l'agenda de l'action, qui s'est déroulée autour de plusieurs temps forts : des plénières d'ouverture et de clôture où des messages forts sur l'importance de la prise en compte de l'eau dans les stratégies de résilience et de lutte contre le changement climatique ont été délivrés. ont été délivrés. Une déclaration a été faite pour soutenir les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau dans le contexte du changement climatique, portée par les alliances mondiales pour l'eau et le climat, avec le soutien actif de la France et de l'Italie,

l'eau dans l'agriculture ou encore la connaissance scientifique de l'eau. Enfin, de nombreux autres événements sur l'eau se sont déroulés, notamment au pavillon français. La France se félicite donc de la mobilisation de tous les acteurs, de tous les élus, des entreprises et des acteurs non étatiques durant la journée de l'eau, qui fait partie aussi, de façon totalement intégrante, des discussions et des résultats de la COP23.

et des actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement à l'échelon européen. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il est parfois